qui allierait écologie et agriculture et qui s'inscrirait dans un plan plus global d'aide et de sauvegarde de la filière betteravière, de soutien à la recherche d'alternatives à ces pesticides nocifs. On nous dit aussi que la dérogation à l'interdiction de l'usage des néonicotinoïdes serait suffisamment encadrée pour ne pas constituer une régression environnementale. Il s'agirait donc d'un choix responsable. Pourtant, il n'en est rien, car, ce qu'illustre ce choix, c'est surtout l'incapacité de l'État et du Gouvernement à prendre la mesure de l'urgence environnementale et à accompagner la transition agroécologique, et ce depuis de trop nombreuses années. La Cour des comptes nous l'a très justement rappelé il y a peu, l'échec des politiques publiques qui se sont succédé depuis plus de dix ans pour atteindre l'objectif d'une véritable transformation des modes de production agricole est sans appel

Comme pour le refus d'encadrer la vente des pesticides ou d'interdire le glyphosate, ce choix n'est rien d'autre que la reprise d'une doctrine d'intervention publique largement dépassée, en lieu et place d'une véritable planification volontariste portée tant par le ministère de l'environnement que par celui de l'agriculture une doctrine de l'ancien monde, qui prétend qu'il est possible de réguler les pesticides, en évaluant le risque substance par substance et en définissant les conditions d'un usage contrôlé, censé apporter une garantie de protection pour la santé humaine et l'environnement. Or, dès 2005, l'INRA insistait sur la méconnaissance des effets des pesticides dans leur ensemble et la nécessité d'inciter les agriculteurs français à une moindre consommation. En 2008, le plan Écophyto se fixait l'objectif de réduire de 50 % la consommation de pesticides agricoles en dix ans. Nous en sommes loin ! C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 1. La

Comme vous l'avez compris, notre groupe reste fermement opposé à ce projet de loi. Réautoriser les néonicotinoïdes pour trois ans, et probablement pour toutes les cultures- il faut arrêter de se mentir, c'est bien de cela qu'il est question dans ce texte -, serait une régression environnementale qui irait à contre-courant de l'histoire. Je tiens à rappeler que cette interdiction n'a pas pris au dépourvu les filières. Je vais évoquer ici quelques dates qui montrent qu'elle est le fruit d'un long cheminement dont l'issue est évidente. Dès les années 1990, suite à leur introduction en Europe puis en France, les néonicotinoïdes ont suscité des inquiétudes quant à leur impact sur l'environnement quant à leur impact sur l'environnement et la biodiversité. Pendant plus de vingt ans, les études scientifiques se sont multipliées pour le démontrer. Le consensus est aujourd'hui total. Dès 2012, l'Anses recommandait d'engager une réévaluation de ces substances au niveau européen, et Stéphane Le Foll interdisait le Cruiser, pesticide utilisant une molécule de cette famille. En 2013, suite aux travaux de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, la Commission européenne décidait un moratoire interdisant trois des cinq substances actives de cette famille d'insecticides.

au 1septembre 2018 pour le principe général d'interdiction et au 1juillet 2020 pour la fin des éventuelles dérogations. Personne ne peut donc dire dans cet hémicycle que cette interdiction était précipitée et a pris de court certaines filières. Je vais vous livrer mon sentiment : dans moins de trois ans, j'en suis convaincu, un nouveau projet de loi sera déposé et prolongera ce même système dérogatoire. En 2016, lors du vote de la loi Biodiversité, nous savons que certaines filières avaient déjà parié sur le fait qu'une loi viendrait détricoter cette interdiction d'ici à 2020,

sur le long terme, ainsi que les risques associés à ces substances pour la santé humaine, ce qui justifie un maintien strict de leur interdiction. Nous sommes en attente de deux avis de l'Anses sur la question des alternatives aux néonicotinoïdes. Nous trouvons d'ailleurs très problématique que les débats aient lieu sans que nous ayons ces éléments. estimé lors de son audition qu'il manquait de données pour établir scientifiquement les impacts agronomiques et économiques des alternatives aux néonicotinoïdes sur les filières et, donc, pour établir clairement la situation d'impasse

en se dotant d'une compétence pour réaliser des analyses socio-économiques. La position de la Commission semble aller dans le sens d'un questionnement sur la légitimité de ces dérogations. Nous le répétons, dans une communication du 1octobre, celle-ci estime que l'utilisation par les États membres des dérogations d'urgence sur les néonicotinoïdes pour la betterave sucrière est problématique. Elle a annoncé qu'elle allait saisir l'EFSA

d'indemnisation, de compensation, de fonds de mutualisation ou encore des aides à l'investissement pour la filière. Quel

un avis défavorable. pour explication de vote. Je souhaite revenir sur les raisons qui poussent l'ensemble des sénateurs Socialistes, Écologistes et Républicains à s'opposer à ce projet de loi. L'Anses définit les néonicotinoïdes comme des substances insecticides dites « systémiques », utilisées en agriculture pour protéger les cultures de ravageurs, mais aussi en tant que biocides ou médicaments vétérinaires. Les néonicotinoïdes font partie des insecticides les plus utilisés en France et les plus vendus dans le monde : ils représenteraient 25 % du marché mondial selon le. L'Anses évalue L'Anses évalue qu'ils constitueraient 34 % du volume total des insecticides utilisés en France en 2016 devant les organophosphorés et les pyréthrinoïdes de synthèse. En somme, il s'agit de produits extrêmement présents en France comme en Europe. Dans le même temps, leur impact sur les insectes, particulièrement sur les pollinisateurs du fait de leurs effets neurotoxiques, n'est plus aujourd'hui à démontrer, tant la littérature scientifique est unanime à ce sujet. L'Union nationale de l'apiculture française, l'UNAF, estime ainsi que 300 000 ruches sont anéanties chaque année à cause des néonicotinoïdes. D'une manière générale, certaines études font une corrélation très claire entre leur autorisation et la disparition de 85 % des populations d'insectes

Mes chers collègues, faut-il rappeler les chiffres alarmants que nous donnait, encore l'année dernière, la plateforme des experts pour la biodiversité et les écosystèmes ? Un million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui en voie d'extinction, et le rythme actuel de disparition des espèces est 100 à 1 000 fois supérieur au taux naturel d'extinction. En cause, l'agriculture intensive, l'urbanisation, la déforestation et le recours croissant à des produits chimiques qui polluent et annihilent toute forme de vie.

Les députés socialistes- je salue ici le travail de Dominique Potier notamment -ont d'ailleurs présenté un plan B, comme « betterave », qui permettrait à la filière de sortir durablement de la crise, sans pour autant maintenir l'usage des néonicotinoïdes. Ce plan repose sur trois piliers. Premier pilier : l'innovation commerciale, en fixant l'objectif pour le sucre français d'atteindre 50 % de produits issus de mentions valorisantes, dont 20 % en agriculture biologique d'ici à 2030. Cette montée en gamme de la filière lui permettrait de se positionner sur des marchés fortement émergents actuellement comme, par exemple, le bio. Deuxième pilier : l'innovation économique et sociale, en structurant la filière, qui souffre d'un manque d'instruments de solidarité, pour la rendre plus résiliente face aux aléas. Cela pourrait passer par la création d'une organisation de producteurs regroupant, par exemple, les quatre régions principales concernées. Le Le pacte de solidarité que nous demandons devra évidemment passer par la compensation des pertes de production subies en 2020 et la mise en place d'un fonds de développement doté de 100 millions d'euros, soit 250 euros par hectare, pour maintenir l'attractivité de la filière et lui permettre de s'orienter vers l'agroécologie. Pour financer ce pacte, nous proposons de créer une taxe exceptionnelle sur le secteur agroalimentaire. Troisième pilier : l'innovation agroécologique, en mettant en oeuvre des pratiques agriculturales vertueuses en termes de génétique végétale, de développement du biocontrôle, d'adaptation des dates de semis, ou encore de la création d'une mosaïque paysagère, et de succession culturale propice à un meilleur équilibre écologique. Vous le constatez, nous ne sommes pas que dans l'opposition : nous faisons également des propositions, même si celles-ci- nous vous l'accordons -nécessitent davantage de mobilisation de tous les acteurs que la simple réintroduction des néonicotinoïdes dans un projet de loi exprès. Merci de conclure, cher collègue La capacité de résilience de notre agriculture est la clé de sa sauvegarde dans toute sa diversité. C'est dans ce sens que nous devons concentrer nos efforts. La parole

sans nuance, donnée à l'économie sur l'environnement. Nous, sénateurs Socialistes, Écologistes et Républicains, ne souhaitons pas opposer ces deux objectifs, car nous pensons que nous pouvons les concilier. Toutefois, le Gouvernement ne paraît pas être sur cette position tant les renoncements semblent se multiplier : hier le glyphosate, aujourd'hui les néonicotinoïdes et, demain, l'amoncellement des vetos sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Les exemples de ces renoncements seraient trop nombreux à citer, mais sachez que les parlementaires que nous sommes y sont confrontés au quotidien sur de nombreux textes. Aujourd'hui, nous parlons des néonicotinoïdes, et je ne peux m'empêcher d'évoquer le tweet du Président de la République du 1septembre 2018, qui se félicitait de leur interdiction : « Notre engagement pour la biodiversité en action : l'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles en vigueur aujourd'hui. » Je pense également à la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, qui doit être bien en peine de justifier les propos qu'elle a tenus en 2016 quand, au moment de l'examen de la loi Biodiversité, elle défendait ardemment cette interdiction, en s'opposant même à l'époque au principe des dérogations.

depuis l'entrée en vigueur de la loi Biodiversité en 2018, les approbations européennes de substances actives se sont très significativement réduites. Pour nous, c'est la preuve que, lorsqu'un pays prend ses responsabilités, il peut ouvrir la voie à une prise de conscience collective, à des changements en profondeur. La France avait fait un grand pas en avant en 2016 ; aujourd'hui, vous nous demandez d'en faire trois en arrière. je vous remercie

un effondrement de la biodiversité et du nombre d'insectes. Pour ceux qui étaient nés dans les années 1970, je vous demande de vous rappeler que, lorsque vous rouliez quelques kilomètres en voiture de nuit, vous reveniez avec un pare-brise moucheté, rempli d'insectes

Je suis désolé de vous dire que le système agricole actuel ne fonctionne pas si bien que cela. Aujourd'hui, on ferme 500 exploitations chaque mois, les agriculteurs ont un taux de suicide bien supérieur à la moyenne française, parce que le libéralisme leur a mis un genou

à cultiver des lentilles vertes du Puy, parce que j'estimais que c'était une valeur pour mon territoire, mais aussi parce qu'il s'agit d'une valeur ajoutée importante pour notre agriculture, pour mon exploitation.

Ce projet de loi ne prévoit pas seulement des dérogations à l'interdiction des néonicotinoïdes : l'article 1 réécrit l'ensemble des dispositions votées dans la loi Biodiversité, au motif qu'elles seraient fragiles juridiquement.

il a fait l'objet d'une décision récente de la Cour de justice de l'Union européenne, en date du 8 octobre 2020, qui, elle, a conforté la solidité juridique de l'interdiction française des néonicotinoïdes au regard de sa procédure de notification.

fragilité juridique de l'interdiction de 2016 à l'égard du droit européen, n'a plus lieu d'être. Je propose donc de revenir à la formulation actuelle de l'alinéa de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, qui pose le principe de l'interdiction des néonicotinoïdes et des substances aux modes d'action identiques, puisque celle-ci est, je le répète, sécurisée juridiquement. Cette réécriture étant inutile et dangereuse, il convient, j'y insiste, de revenir à la formulation du principe d'interdiction tel que proposé en 2016.

qui, de l'aveu de tous, présente de forts risques d'inconstitutionnalité pour cause de rupture d'égalité devant la loi. Son introduction à l'Assemblée nationale est purement cosmétique : nous savons bien que, ce que vous permettez aujourd'hui aux betteraviers, vous le permettrez demain à d'autres. Il n'a d'ailleurs pas fallu attendre longtemps pour que d'autres filières demandent à bénéficier de la dérogation. Dès le début du mois d'août, la filière maïs s'est positionnée. Aujourd'hui, celle de la noisette fait de même. Vous avez même eu des demandes directement en séance, il me semble, Nous pensons que l'article 2 n'a quasiment aucune chance de figurer dans la loi qui sera promulguée. Avec cet amendement, nous tenons à mettre tous ceux qui soutiennent ce projet de loi devant leurs responsabilités en mettant fin à ce jeu de dupes.

Ce que la France ne produira plus, elle devra l'importer, c'est-à-dire faire venir des produits qui sont eux-mêmes traités par des produits phytopharmaceutiques que l'on interdit sur notre territoire. Ce constat vaut en particulier pour des productions comme celle de la noisette. En France, nous consommons 25 000 tonnes de noisettes par an ; nous en produisons 11 000 tonnes. Jusqu'à cette année, les producteurs de noisettes disposaient d'un traitement néonicotinoïdes par dérogation. Sans celui-ci, et en attendant des solutions alternatives plus écologiques, souhaitées par tous, mais qui tardent à venir, les agriculteurs ne disposeront plus de solution satisfaisante pour lutter efficacement contre le balanin,

à pouvoir les aider à trouver des alternatives, alors même qu'elles n'ont pas des capacités de recherche extrêmement importantes. Aussi, je vous repose la question de ce que vous prévoyez pour elles. Néanmoins, mon cher collègue, l'amendement qui nous est présenté ne peut trouver sa place dans ce texte.

cette dérogation doit se limiter à la betterave sucrière, en raison des deux spécificités que j'ai évoquées : moindre impact sur les pollinisateurs que d'autres cultures, du fait d'un caractère non mellifère de la plante, c'est-à-dire qu'elle est récoltée avant culture, ce qui n'est pas le cas, par essence, avec le noisetier ; dépendance à l'appareil de production en aval, qui peut fermer en l'espace d'une seule saison. S'agissant des maladies liées à la noisette, il y a

Sauf urgence, bien entendu, le ministre pourra suspendre une autorisation de mise sur le marché ou interdire l'utilisation d'un produit après un bilan de l'Anses mesurant les bénéfices et les risques liés à l'utilisation de produits de substitution ou de méthodes alternatives, qu'elles soient chimiques, de biocontrôle, qu'elles relèvent de la génétique ou de l'agronomie. Si un produit n'a pas d'alternative, le Gouvernement aura ainsi toutes les cartes en main pour décider ou pas une interdiction. De même, l'Anses, comme aujourd'hui, tiendra compte dans ses décisions de retrait d'AMM, des risques liés aux alternatives proposées ou, bien sûr, de l'absence d'alternative. C'est un amendement de bon sens, qui rappelle qu'il est nécessaire d'étudier l'impact d'une interdiction avant de la décider, sauf, évidemment, en cas d'extrême urgence. Nous nous battons tous les jours pour demander au Gouvernement une amélioration des études d'impact accompagnant les projets de loi, afin de prendre des décisions plus raisonnées. Je sais que c'est un sujet qui tient à coeur à de nombreux sénateurs ici présents, notamment MM. Montaugé et Cabanel. Par cet amendement, nous proposons, dans le même esprit, d'améliorer l'étude d'impact préalablement établie à l'interdiction d'un produit afin de ne pas laisser des agriculteurs sans solution, car nous avons vu ce que cela peut donner.

je m'intéresse de près à la question des mines industrielles, notamment en Guyane, et à la cyanuration, qui est destructrice pour l'environnement et les peuples autochtones. Aujourd'hui, il existe des alternatives, il en existe même trois,

en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées imposées par cette même réglementation. « L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa. » Force est de constater que ce n'est pas encore le cas. Comme l'a rappelé Laurent Duplomb dans un rapport d'information, les importations de denrées alimentaires prennent une place de plus en plus importante dans la consommation des Français. Or rien aujourd'hui ne garantit qu'elles respectent les normes de production minimales imposées à nos propres agriculteurs, notamment en matière de produits phytopharmaceutiques. En outre, les accords de libre-échange accentuent ce phénomène, les négociations à l'échelon européen se poursuivant avec de nombreux pays, sans que ces accords prévoient des clauses suffisamment protectrices pour nos agriculteurs et nos consommateurs.

La souveraineté alimentaire passe donc par là. La loi consolidera peut-être l'interdiction des néonicotinoïdes en France, mais rien n'interdit que ces substances soient utilisées dans les produits importés, d'ici d'ici à 2023, quand les dérogations prendront fin, d'autant plus si les alternatives ne sont pas suffisamment efficaces. Sera-t-il acceptable de laisser s'installer une concurrence déloyale avec les pays européens et les pays extraeuropéens qui utiliseront ces produits ? Dès lors, cet amendement vise, dans le strict respect du droit européen, à donner aux ministres de l'agriculture et de la consommation le pouvoir de prendre des mesures conservatoires, lorsqu'il est constaté que cette concurrence déloyale est établie. Cela inclut les concurrences déloyales aux produits phytopharmaceutiques posant un risque pour l'environnement ou la santé, mais aussi les médicaments vétérinaires, les aliments pour animaux non autorisés à l'échelon européen et les produits ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité nécessaires. Quel est l'avis du Gouvernement

loin en prévoyant que le ministre de l'agriculture et le ministre de la consommation, c'est-à-dire Bercy, puissent prendre la décision d'interdire la vente sur le marché de substances qui ne respectent pas les mêmes règles, et de l'article 53 du règlement européen : « Lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine communautaire ou importés d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement

non pas dans la politique agricole commune, mais dans les politiques commerciales et dans les accords de libre-échange. À partir du moment où l'on se met tous d'accord sur un socle environnemental contraignant à tous les États membres,

sans jamais nous consulter. Au moins, là, ils auront une feuille de route

M. le ministre. Il me revient la lourde tâche de défendre une position face à un consensus absolu, que je respecte et que je comprends

En application de l'article 43, alinéa 4, du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération de l'article 1.